L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à Mme Marion Canalès, Dans un contexte de réchauffement climatique ayant pour conséquence directe une multiplication des périodes de stress hydrique à l’échelon national et une raréfaction de cette ressource essentielle, une réflexion globale doit être menée avec tous les acteurs concernés autour des enjeux de gestion, de préservation, mais aussi de financement des politiques dédiées à l’eau. Il s’agit de penser global et d’agir local. C’est ainsi qu’en conclusion des Assises de l’eau organisées en 2019 a été annoncée une réforme des redevances des agences de l’eau.

pour le prélèvement de l’eau due par les agriculteurs irrigants, afin de tendre vers un système plus sobre, plus résilient et plus concerté. Ensuite a été prévue une augmentation de 20 % de la redevance pour pollutions diffuses Cette taxe, perçue sur les ventes de pesticides, finance directement les programmes de traitement des eaux des agences de l’eau, ainsi que les mesures du plan Écophyto, qui prévoit de réduire de moitié l’usage des pesticides d’ici à 2030. Cette mesure n’a pas été tout à fait à la hauteur. Pourtant, il serait moins coûteux de lutter contre la pollution avant qu’elle ne survienne, plutôt que de traiter l’eau traiter l’eau pour l’alimentation en eau potable. Cela représente une diminution de 47 millions d’euros pour le financement d’un plan Eau qui prévoit de doter les agences de l’eau de 475 millions d’euros supplémentaires chaque année. Cette hausse annuelle du financement se révèle nécessaire au regard des enjeux, mais aussi des efforts très importants que doivent supporter les collectivités territoriales pour le traitement de cette ressource rare. Monsieur le ministre, quelles mesures comptez vous prendre pour tenir les engagements financiers annoncés ? Selon vous, qui assumera les deltas et compensera les millions d’euros qui manqueront, afin de garantir la mise en œuvre pleine et entière du plan Eau ? La parole

Ainsi, les redevances qui s’appliquent aux usagers raccordés aux réseaux d’eau potable et d’assainissement sont réformées en profondeur afin de donner aux instances des agences de l’eau

à l’exception des éleveurs pour l’abreuvement des animaux, seront également assujettis sur des bases identiques. La redevance de prélèvement est également modifiée en profondeur, avec un relèvement des taux plafonds

Ces taux planchers ont pour conséquence une augmentation des rendements de 120 millions d’euros – 100 millions d’euros pour l’énergie nucléaire et 20 millions d’euros pour l’industrie. sont nuls à ce stade pour l’irrigation gravitaire et non gravitaire, avec la perspective de déterminer une trajectoire pluriannuelle d’évolution de ces planchers à compter de l’an prochain. Par ailleurs, des dispositions sont introduites pour inciter au comptage de l’eau, avec la majoration de la redevance en cas d’absence ou de défaillance du système de comptage et l’augmentation progressive du forfait

La parole est à M. Jean Michel Arnaud,

pour améliorer sa protection et conforter un projet de territoire durable au service de la qualité de vie des habitants. Ces principes génériques permettront d’ouvrir les espaces. Il va de soi que les parlementaires seront étroitement associés

Lundi prochain, nous serons un certain nombre de parlementaires à assister au lancement de la COP Région Île de France, aux côtés du Gouvernement. L’objectif de cette conférence régionale des parties est de travailler collectivement pour permettre à la région d’atteindre ses objectifs

avance à grand bruit avec le démarrage des travaux préparatoires, notamment de nombreux défrichements, malgré l’opposition unanime des associations locales et des populations qui en subiront les nuisances. Ce projet vieux de 40 ans, fruit d’une vision obsolète de l’aménagement, induira une hausse du trafic de 114 % dans une boucle enclavée de la Seine, entraînera nuisances et pollutions, affectera la santé des riverains et provoquera la destruction d’écosystèmes précieux dans mon département – sans parler des coûts d’entretien dans les années à venir, dont on sait aujourd’hui qu’ils seront difficilement supportables. Pour quels bénéfices ? Monsieur le ministre, que compte faire concrètement le Gouvernement face à ce projet, source d’une profonde incompréhension chez une grande partie de nos concitoyens, tant il entre en contradiction avec les engagements et les objectifs que s’est fixés la France à l’heure du tournant écologique ? La parole est

aux « circonstances nouvelles » intervenues au cours de l’exécution du contrat. Il en résulte des hausses très importantes des primes d’assurance et du montant des franchises, mais surtout de nombreux refus d’assurer. lors du renouvellement de leur marché, de nombreuses communes n’ont reçu aucune candidature à leur appel d’offres. L’augmentation des épisodes climatiques violents fait peser des risques accrus sur les communes, notamment rurales. La question de leur couverture, même partielle,

Nous sommes absolument déterminés à accompagner les élus locaux, non pas seulement parce qu’ils participent à l’action publique, mais parce qu’ils constituent le levier essentiel, au quotidien, des politiques destinées à nos concitoyens. Nous agissons à court terme. Avec l’appui de la direction générale du Trésor, nous avons étendu la compétence du médiateur de l’assurance

L’une des solutions pour répondre à cette crise du logement consiste à élargir la segmentation du parcours résidentiel. Les font partie intégrante de cette nouvelle segmentation, comme l’ensemble des habitats légers. acquisition ne peut être financée que par des prêts à la consommation dont la durée de remboursement et les taux sont moins intéressants que ceux des crédits immobiliers classiques. Ces petites maisons disposent pourtant de nombreux avantages : coût faible, délai de construction rapide, très bonne performance énergétique. Elles représentent une véritable solution de logement de transition pour une large frange de la population, notamment les saisonniers, les étudiants et les jeunes couples d’actifs. À l’heure actuelle, l’impossibilité d’avoir recours à un crédit immobilier pour les financer freine leur développement et empêche l’amélioration de cette segmentation du parcours résidentiel, qui devient de plus en plus nécessaire. monsieur le ministre, je vous demande d’étudier des formes de financement pérenne pour ce type de logement.

certains jeunes en alternance renoncent à suivre leur formation théorique en CFA et se consacrent uniquement à l’acquisition des savoir faire en entreprise. Ce renoncement peut être lié à un manque de motivation pour la formation dans laquelle ils se sont engagés. Il peut également être la conséquence de difficultés particulières en matière d’acquisition des connaissances : le jeune estime ne pas avoir le niveau scolaire suffisant et baisse rapidement les bras. En entreprise, en revanche, ces jeunes sont souvent appréciés pour leur motivation et la qualité de leur travail et peuvent être incités à quitter l’alternance pour conclure un CDI. Chacun est gagnant dans cette relation : l’entreprise, d’une part, qui attire une main d’œuvre parfois excellente dans des secteurs d’activité faisant face à de sérieuses difficultés de recrutement ; le jeune, d’autre part, qui perçoit une rémunération et ne reste pas inactif. cette situation se révèle finalement pénalisante pour les jeunes concernés, qui perdent le bénéfice de leur formation et se retrouvent sans diplôme au terme de leur parcours en CFA. En outre, l’absence de diplôme leur interdira d’évoluer ultérieurement dans le domaine professionnel. J’ajoute que le CFA ne dispose d’aucun moyen d’action propre permettant d’influer sur la décision des alternants de céder à une proposition d’embauche avant d’avoir finalisé leur cursus. Aussi, monsieur le ministre, je souhaite connaître vos propositions en faveur du renforcement des dispositifs d’accompagnement des élèves et de la prévention du décrochage. La parole est à M. le ministre.

permettre aux jeunes peu ou pas qualifiés de renforcer leurs savoirs fondamentaux et de mieux appréhender les codes de l’entreprise, afin de préparer efficacement l’entrée en apprentissage et de sécuriser un contrat. C’est aussi un moyen de leur faire savoir exactement à quoi ils doivent s’attendre et de leur éviter de bifurquer.

Force est de constater que, depuis 2006, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) n’a quasiment pas fait évoluer le montant alloué aux résidents des maisons d’accueil spécialisées (MAS) accueillis en Belgique. le coût de la prise en charge des résidents n’a fait qu’augmenter, en raison non seulement de la croissance des salaires du personnel encadrant, mais également de l’inflation du coût des biens et des services. Les institutions belges sont désormais à l’os.

De plus, il est à noter que la CNSA a régulièrement revalorisé le montant alloué pour les résidents des MAS accompagnés en France, au point que les résidents français hébergés en Belgique ont un forfait journalier inférieur de plus de 20 % avec la médiane des Français hébergés en France ! Monsieur le ministre, pourriez vous clarifier la position de la CNSA sur cette discrimination ? Serait il envisageable que le prix de journée octroyé par la CNSA aux résidents des MAS séjournant en Belgique soit aligné sur la médiane de celui des résidents des MAS accueillis en France ? Enfin, serait il possible que les établissements belges bénéficient d’un mécanisme de revalorisation annuelle du prix de journée, à l’instar des établissements français ? La parole

uniquement dans le nord et le nord est du pays, de manière à prévenir ces départs non souhaités. Telle est notre orientation principale.

Ils créent et nourrissent le lien social, mettent en œuvre des politiques publiques, participent à l’amélioration des conditions de vie, proposent des activités sociales, culturelles et familiales et contribuent à l’attractivité de nos territoires. Dans le Cantal, près de 8 000 usagers sont ainsi accueillis dans des centres animés par plus de 125 associations et employant 400 salariés permanents.

était nécessaire, il entraîne une hausse significative de la masse salariale qui s’ajoute à l’inflation actuelle et qui aura des répercussions notables sur les budgets de ces structures. Cette augmentation fait peser des interrogations sur l’avenir même de ces centres sociaux associatifs. Des choix risquent d’être faits, au détriment des habitants de nos territoires, et, au final, peut être même des salariés, faute de moyens.

J’appelle votre attention sur le fait que l’augmentation de la masse salariale pour les structures couvertes par d’autres conventions collectives est, non pas de 8 %, mais de 4 %.

des solidarités. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger aujourd’hui sur les revendications relatives à l’application de l’augmentation de la valeur du point des personnels des réseaux associatifs d’aide à la personne

par des trottinettes électriques et autres engins motorisés individuels. Ce bilan, déjà inquiétant, est de plus en très forte hausse chaque année, conséquence directe de l’explosion de ces circulations douces. Chaque mois, chaque semaine, la presse relate de nouveaux accidents graves. – c’est peu de le dire – est devenu anxiogène. La politique de la municipalité aggrave les embouteillages et les mobilités douces causent la frayeur des poussettes, quand elles ne renversent pas des passants, qui sont parfois des âgées. S’il est essentiel d’encourager les nouvelles mobilités, il faut également réglementer leur usage. Or le partage de l’espace public, mal pensé et plus mal exécuté encore par la majorité municipale, entraîne des conflits entre les usagers, notamment dans les zones piétonnes que crée la Ville de Paris.

Hélas, cela n’a pas permis de sécuriser la circulation. Cette interdiction n’a même servi à rien, puisqu’elle s’est traduite par un report vers l’achat ou la location de trottinettes.

Pouvez vous donc nous préciser, monsieur le ministre, quelles politiques vous comptez mettre en place pour faire baisser le nombre d’accidents et d’incivilités sur la voie publique à Paris ? La parole

Le préfet de police a pour sa part des compétences d’attribution sur le fondement de la sécurité des personnes et des biens et de la protection des institutions, en particulier pour les sites sensibles. Il dispose également d’un rôle prescriptif pour les aménagements

une hausse de 11,4 %, soit près de 5 000 verbalisations, contre 4 400 l’année précédente. De manière plus générale, la politique de sécurité routière qui est menée par la préfecture de police s’inscrit dans le prolongement du document général d’orientation

dans ce DGO, en 2024, la préfecture de police sera plus particulièrement attentive aux infractions commises par les conducteurs d’engins de déplacement de mobilité douce, en ciblant à la fois les infractions relatives à la signalisation, au non respect des passages piétons et des feux tricolores qui, dans beaucoup de cas, provoquent ou augmentent ce nombre d’accidents.

Ce format maximal est il arrêté, définitif, réalisable et tenable dans la durée pour nos forces armées ? L’incertitude actuelle quant à l’ampleur exacte de la mobilisation et le manque d’informations précises posent des défis non seulement opérationnels, mais aussi logistiques et humains. La gestion du personnel, la préparation des infrastructures et le soutien logistique nécessitent une attention particulière. Ces préoccupations s’étendent aux conditions d’hébergement des soldats, aux indemnités allouées et à l’organisation des permissions. Il est essentiel que nos militaires mobilisés sur le territoire national bénéficient de conditions de vie et de travail décentes, que leur rôle soit valorisé au même titre que celui de leurs camarades des forces de sécurité intérieures, gendarmes, Comment le ministère compte t il garantir des conditions d’accueil dignes, une rémunération adéquate et une gestion humaine des permissions pour ces hommes et ces femmes dévoués à la sécurité de notre Nation ? De plus, quelle stratégie est envisagée pour minimiser les conséquences de cette mobilisation sur les missions et les formations programmées ? Comment nous assurerons nous que cette opération cruciale pour la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques ne se fasse pas au détriment de la préparation et de la disponibilité opérationnelle de nos forces pour d’autres engagements essentiels

Le ministère de l’intérieur et des outre mer, dont c’est la responsabilité, planifie et prépare depuis de nombreux mois la sécurisation de ces Jeux qui interviendront dans un contexte stratégique très incertain compte tenu de l’état du monde et de la situation géopolitique. La nature des La nature des menaces auxquelles notre pays doit faire face et l’ampleur des moyens nécessaires pour s’y opposer imposent que les armées se joignent à cet effort en apportant leur appui au ministère de l’intérieur. Cet appui sera réalisé dans les conditions prévues par le code de la défense, c’est à dire sur réquisition et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme militarisé, pour assurer les postures permanentes de sauvegarde maritime et de sûreté aérienne.

concerne l’ensemble du territoire national, tant l’Hexagone que les outre mer, avec un engagement dès le printemps, dès l’arrivée de la flamme olympique et jusqu’à la fin des jeux Paralympiques au mois

puissent être accompagnés au mieux. En ce qui concerne enfin la rémunération, les militaires qui seront engagés dans le cadre de l’opération Sentinelle bénéficieront à ce titre de l’indemnité d’absence opérationnelle au taux maximum.

des échéances prévues par les textes applicables, notamment les délais d’inscription, pour que chacun ait le temps. Comme vous le relevez, madame la sénatrice, lors des élections de 2019, la charge de travail, induite notamment par les consultations des différents acteurs impliqués, a eu pour conséquence un glissement de calendrier d’un mois, amenuisant mécaniquement la période d’inscription sur les listes électorales. Dans le cadre de la préparation du prochain scrutin, les préfets feront afficher dès que possible, mais au plus tard le 1 juillet 2024, les avis annonçant l’établissement des listes électorales pour l’ensemble des collèges d’électeurs. Ainsi les intéressés pourront ils faire connaître leur demande d’inscription sur les listes électorales durant une période minimale de deux mois et demi.

et numérique. Monsieur le ministre, ma question porte sur la situation du marché du crédit immobilier. Depuis plusieurs mois, le secteur immobilier subit une crise d’ampleur qui touche à la fois tout Français souhaitant se loger et tous les secteurs qui dépendent du marché du crédit immobilier. Cela affecte également les collectivités territoriales, qui ont vu baisser leurs recettes liées aux droits de mutation. Si cette crise résulte en grande partie de la hausse des taux d’intérêt, un facteur aggrave la crise actuelle, à savoir les nouveaux critères décidés par le Haut Conseil de stabilité financière. Ces critères obligatoires plafonnent le taux d’endettement à 35 % sans tenir compte du reste à vivre des ménages. La durée d’emprunt ne peut, quant à elle, excéder vingt cinq ans pour l’ancien et vingt sept ans pour le neuf. Les principales conséquences de cette nouvelle réglementation sont les refus de plus en plus nombreux de crédits et des allongements de durée non nécessaires et coûteux pour les emprunteurs. Les règles du Haut Conseil de stabilité financière bloquent des Français pourtant solvables et finançables. Face à la crise actuelle et à ces nouvelles règles contraignantes, c’est tout le marché immobilier qui est fragilisé. Les acteurs du marché immobilier demandent plus de flexibilité dans l’application des règles établies par le Haut Conseil de stabilité financière, notamment une meilleure prise en compte du reste à vivre des foyers. Une telle mesure ne coûterait rien aux finances publiques. Monsieur le ministre, vous paraît il envisageable de modifier la réglementation en vigueur pour rendre plus flexibles les règles du Haut Conseil de stabilité financière et ainsi relancer le secteur de l’immobilier qui en a tant besoin ? La parole est à M. le ministre.

monétaire. La baisse de la demande des ménages est en effet causée par la hausse rapide des taux d’intérêt immobiliers et constitue la raison principale de la baisse de production de crédit. Récemment, les taux d’intérêt tendent toutefois vers une stabilisation qui pourrait ralentir la dégradation des conditions de financement.

de ne pas freiner l’offre de crédit, tout en respectant les grands principes. Premièrement, la marge de flexibilité de la mesure a été élargie s’agissant de la partie libre d’utilisation, par exemple pour soutenir l’investissement locatif. Deuxièmement, le respect de la marge de flexibilité sera désormais apprécié par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur trois trimestres glissants, ce qui permet aux banques un ajustement plus souple, notamment pour tenir compte des pics de saisonnalité. Troisièmement, les prêts relais sont désormais exclus du calcul du taux d’effort, sous condition de quotités de financement de 80 % au maximum, afin de fluidifier le marché. la possibilité d’allonger la maturité des prêts avec un différé d’amortissement est facilitée dans le cas de la construction d’un logement neuf ou dans le cas de travaux dont le montant s’élève à moins de 10 % du coût total de l’opération. Le Gouvernement soutient enfin la mise en place par la Fédération bancaire française d’un dispositif offrant la possibilité d’un réexamen pour les ménages solvables dont la demande de crédit immobilier aurait été refusée.

un choix qui profiterait à Transavia, filiale du groupe. Ce transfert aurait pour conséquence le départ de 600 à 1 000 emplois d’Orly, sans compter les emplois induits, estimés à 1 pour 5. Cela conduirait – permettez moi l’expression, monsieur le ministre – à un véritable « désarmement économique » du Val de Marne et du sud francilien. L’État est le premier actionnaire d’Air France. Il lui alloue en outre des subventions au titre de sa mission de continuité territoriale. Pourtant, pas une seule fois le Gouvernement ne s’est exprimé. aéroport français et douzième aéroport européen, Orly est l’aéroport le plus dynamique d’Île de France et la passerelle avec les outre mer. Cette dynamique fragile repose sur une diversité d’activités : présence d’Air France, industries à proximité, croissance des vols à bas coût et développement des longs courriers. L’argument des économies après regroupement d’activité ne tient pas. Le potentiel d’Orly continue de s’accroître. Des compagnies privées sans mission de service public sont avides de récupérer des lignes, y compris pour la Corse. J’en viens donc à mes deux questions, monsieur le ministre. Le Gouvernement entend il maintenir les emplois et les lignes d’Air France à Orly ? Quelle est la vision stratégique du Gouvernement pour l’avenir de l’aéroport d’Orly ? La monsieur le ministre. d’abord sur un constat simple : la demande des vols sur le réseau national s’est effondrée depuis la crise sanitaire, du fait principalement de l’attractivité du train et du développement du travail en distanciel, ce qui entraîne des pertes importantes pour Air France, alors même qu’Orly,

et dont le premier exemplaire été livré à Orly il y a tout juste une semaine. Enfin, pour ce qui est de la desserte du territoire, la direction d’Air France s’est engagée à maintenir 90 % de l’offre existante sur le réseau national et le groupe continue d’avoir des discussions avec les élus locaux

et numérique. Monsieur le ministre, en 2019, le groupe russe Novatek annonçait le lancement du projet Arctic LNG 2 de gaz naturel liquéfié en Arctique. Ce chantier, très stratégique pour la Russie, devait lui permettre de produire et d’exporter 20 millions de tonnes de gaz liquéfié par an vers l’Europe et l’Asie. La filiale française était liée contractuellement au groupe russe à hauteur de 7 milliards d’euros pour assurer l’ingénierie et la construction du projet. La guerre en Ukraine a entraîné la mise en application de sanctions à l’échelon européen, interdisant « explicitement les exportations vers la Russie de produits et de technologies utilisés dans la liquéfaction de gaz naturel, et proscrit toute assistance technique, financière ou logistique à leur utilisation ». À la suite d’une enquête du journal, de sérieux doutes sont apparus sur les activités du groupe Technip Energies en Russie. En effet, il semblerait que la société soit parvenue à retarder sa sortie du mégaprojet, notamment avec la poursuite de la livraison de pièces jusqu’au mois d’octobre 2022 et le transfert d’entités

pour qu’ils soutiennent Technip Energies dans le cadre de sa sortie ordonnée du projet. Monsieur le ministre, étiez vous au courant d’un quelconque contournement des sanctions par le groupe Technip Energies pour répondre aux exigences contractuelles du client russe Novatek ? Cette potentielle violation du régime de sanctions fera t elle l’objet d’une enquête ? À la suite des révélations du journal, avez vous exigé la liste des composants de tous les équipements livrés par Technip Energies après la mise en application des sanctions européennes ?

les sanctions européennes contre la Russie comprennent une interdiction de fourniture de biens utilisés dans le raffinage et la liquéfaction de gaz naturel, conformément au règlement de l’Union européenne n° 833/2014. Ce règlement est d’application directe et il est de la responsabilité des entreprises concernées de s’y conformer, en sollicitant les autorisations nécessaires auprès du service des biens à double usage et de la direction générale du Trésor. Vous évoquez des échanges entre le groupe Technip Energies et les services de l’État. L’administration de mon collègue Bruno Le Maire se tient en effet à la disposition de toutes les entreprises françaises sur ce sujet, y compris pour les aider dans leurs démarches de retrait du marché russe.

Le recours accru à la sous traitance pour les raccordements de nouveaux clients a endommagé le réseau, de sorte que des remises en état sont nécessaires. Reste que les différents opérateurs commerciaux La confusion totale qui découle de cette situation a durablement dégradé le réseau de fibre optique de ces communes, ce qui n’est pas sans conséquence sur la qualité de vie de leurs habitants. Cela contraste avec le déploiement du programme

quelles mesures envisagez vous de prendre pour mettre fin à l’anarchie entre les différentes parties prenantes du dossier et quels moyens allez vous engager pour que toutes les communes qui connaissent ces difficultés retrouvent un réseau de fibre optique digne de ce nom ? La parole

les opérateurs commerciaux de leurs plannings d’intervention et grâce à la réalisation de comptes rendus d’intervention permettant le contrôle mutuel entre opérateurs, pour éviter que chacun échappe à sa propre responsabilité. Le troisième axe concerne la reprise des infrastructures dégradées, que ce soit au niveau des points de mutualisation ou des réseaux vieillissants ou mal dimensionnés qui nécessitent une reprise globale de l’infrastructure. Plusieurs opérateurs ont déjà notifié un plan de reprise de 1 000 points de mutualisation à l’Arcep, ce qui correspond à 450 000 locaux. D’autres reprises sont à prévoir.

Interpellée par des élus de mon territoire qui sont concernés par la construction de deux nouveaux EPR2 () à Penly – le début des travaux est prévu en 2027 –, je me fais le relais d’un sentiment d’incompréhension légitime vis à vis de la redistribution fiscale de l’Ifer.

en l’espèce la communauté de communes de Falaises du Talou. Cette exclusivité est prévue par le code général des impôts et s’applique à d’autres cas d’installation de production d’électricité. Le sénateur Hervé Maurey l’a déjà souligné dans sa question écrite du 19 décembre 2019 : cette privation des bénéfices fiscaux légitimes liés à ces installations est

L’éducation nationale souffre, c’est indéniable, et nos enfants sont les premières victimes. Si certaines familles font le choix de l’enseignement privé comme solution de remplacement, tout le monde n’y a pas forcément accès, quelles qu’en soient les raisons.

Ainsi, le montant de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves a été augmenté. La prime d’attractivité a été étendue et revalorisée pour les professeurs stagiaires. Par ailleurs, les professeurs effectuant des missions complémentaires sur la base du volontariat peuvent

les professeurs apprennent à nos enfants et à nos jeunes des savoirs essentiels. Qu’ils exercent dans le privé ou dans le public, ils rendent le même service public d’éducation et de formation des citoyens de demain. des disparités existent entre les professeurs exerçant dans le public et les professeurs des établissements privés sous contrat. En effet, ces derniers se retrouvent écartés des concours de recrutement des professeurs agrégés (Prag) et des professeurs certifiés Aujourd’hui, seuls les professeurs titulaires de la fonction publique peuvent être affectés comme enseignants dans le supérieur. Pour y prétendre, les enseignants du privé ont deux options options : être lauréats d’un concours de l’enseignement public ou demander leur intégration dans le corps des professeurs agrégés ou des professeurs certifiés. Ces étapes supplémentaires sont vécues comme une injustice pour les professeurs des établissements privés sous contrat. Certains interviennent régulièrement dans le supérieur, mais seulement en tant que vacataires. Ils sont en effet privés du statut de titulaire.

je vous remercie public, mais ne sont pas fonctionnaires, comme vous l’avez rappelé. En application de l’article L. 442 5 du code de l’éducation, ils sont détenteurs d’un contrat pour enseigner en classe, fonction pour laquelle ils sont employés et rémunérés par l’État. S’ils bénéficient, en application

en application de l’article L. 513 1 du code général de la fonction publique, car cette position administrative est réservée aux seuls fonctionnaires. Le recrutement de professeurs agrégés et de professeurs certifiés dans l’enseignement supérieur se fait par la voie du détachement ou de l’affectation des membres des corps des professeurs titulaires de l’enseignement public. À ce jour, cette voie est donc fermée aux enseignants du privé. Toutefois, les maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé, lauréats d’un concours de l’enseignement public, qui avaient opté pour leur maintien dans l’enseignement privé, peuvent accéder au recrutement de professeurs agrégés ou de professeurs certifiés affectés dans l’enseignement supérieur en demandant leur intégration dans le corps des personnels enseignants du second degré auquel ce concours donne accès. Par ailleurs et pour prolonger la question que vous posez, une concertation est en cours avec les organisations syndicales des enseignants du privé pour réfléchir aux mobilités nouvelles qui pourraient leur être proposées afin de mieux répondre à leurs attentes. La

et Paralympiques. Monsieur le ministre, comme tous les établissements recevant du public, les écoles doivent respecter des normes relatives à la prévention des incendies. Ainsi, les directeurs d’école doivent être formés à la manipulation des extincteurs.

Ce défaut avait déjà été signalé lors des visites précédentes en 2010, 2015 et 2018. Tenu informé de l’avis défavorable à la poursuite de l’activité d’accueil du public qui s’est ensuivi, le maire s’est vu

plusieurs cas dans la Drôme, dans la Sarthe et ailleurs ont été signalés par des parlementaires. Ce constat est d’autant plus alarmant au vu de l’âge des élèves en école maternelle et primaire. Dans ce contexte, je vous remercie de bien vouloir m’indiquer quelles sont les mesures envisagées pour assurer cette formation indispensable à la sécurité des élèves et du personnel de ces établissements.

Concernant la prévention du risque incendie, les académies sont chargées de mettre en œuvre l’ensemble des mesures prévues, d’une part, par la réglementation des établissements recevant du public, d’autre part, par le code du travail. Ces mesures comprennent la formation du personnel au risque incendie, à la manipulation des extincteurs, au déclenchement de l’alarme et, bien évidemment, à l’évacuation.

Ainsi, dans les orientations stratégiques ministérielles (OSM) en matière de politique de prévention des risques professionnels portant sur l’année 2023, publiées au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 18 du 4 mai 2023, les académies sont invitées à porter une attention particulière à l’évaluation et à la prévention des risques bâtimentaires, notamment le risque incendie.

à la manipulation des extincteurs. Le ministère restera attentif à la mise en œuvre des formations incendie dans les académies et au suivi de la levée des prescriptions formulées par les commissions consultatives

Devant les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie, le Président de la République s’est engagé à bâtir un projet de loi avant la fin de l’été 2023. Au début du mois de décembre dernier, le Gouvernement a annoncé que ce projet de loi sur le modèle français de la fin de vie

La question de la fin de vie mérite d’être débattue au Parlement au nom de nos malades français atteints de maladies graves et souvent incurables. J’ai été particulièrement sensible au témoignage d’un père de famille de mon département qui souffre de la maladie de Charcot. Cette maladie touche environ 9 000 personnes en France et 1 500 nouveaux cas sont déclarés chaque année, soit près de 5 nouveaux cas par jour. Après l’apparition des premiers symptômes, l’espérance de vie des malades est en moyenne de deux à cinq ans.

contrairement à d’autres maladies dégénératives, avec la maladie de Charcot, vos capacités cognitives ne sont pas touchées, vous permettant ainsi de profiter pleinement de votre propre déchéance

Sur la question de la fin de vie, depuis plusieurs années, les mentalités et les attentes de notre société évoluent. Vous l’avez souligné dans votre propos. L’allongement de l’espérance de vie, le nombre croissant de maladies – vous en avez cité certaines –, la dépendance et parfois la souffrance des malades soulèvent de nouvelles questions auxquelles il nous faut répondre. S’il est indispensable d’œuvrer au renforcement de la prise en charge de la souffrance, notamment en soins palliatifs, nous ne pouvons pas ignorer la détresse de ceux qui demandent une aide active à la fin de vie. Conformément aux engagements qu’il a pris, le Président de la République a souhaité que le Gouvernement lui présente un projet de loi sur l’accompagnement de la fin de vie. La ministre du travail, de la santé et des solidarités présentera dans les prochaines semaines une stratégie décennale pour accélérer le développement des soins palliatifs et pour améliorer le droit des patients et la protection des personnes. Celle ci comprendra notamment une réflexion sur l’accompagnement du deuil, sur les directives anticipées et sur l’accompagnement des aidants dans cette période difficile qu’est la fin de vie. volet concernera l’introduction dans notre loi d’une aide active à mourir. Il nous faudra légiférer avec précaution et prudence, dans le dialogue et le respect des professionnels de santé et des familles. Le travail de coconstruction que nous avons engagé sur ce sujet avec le Parlement depuis plus d’un an permettra de trouver un chemin – j’en suis certaine. La ministre du travail, de la santé et des solidarités ainsi que la ministre des relations avec le Parlement détailleront dans les semaines qui viennent le calendrier précis de l’examen parlementaire.

qui, ne pouvant être présente ce matin, m’a chargée de vous répondre en son nom. Le Gouvernement est engagé dans l’amélioration et la protection de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse. Il partage pleinement l’objectif de diversifier les professionnels susceptibles de réaliser des IVG

faisant suite à une expérimentation porteuse de nombreux enseignements, a donné lieu à une large concertation avec les principaux acteurs impliqués, évoquant notamment la question du terme possible de réalisation des IVG dans le cadre de cette pratique.

Ces conditions préexistaient dans le cadre expérimental et elles ont montré toute leur utilité. Cette extension des compétences des sages femmes est une avancée importante pour l’accès à l’IVG de toutes les femmes, en particulier dans des territoires où les contraintes liées à la démographie des professionnels de santé fragilisent celui Le Gouvernement sera particulièrement attentif à sa mise en place concrète dans le plus grand nombre possible d’établissements de santé sur le territoire. C’est également une mesure importante en faveur de la diversification des compétences des sages femmes et de l’attractivité de leur métier dans le cadre hospitalier.

Les stades et les fan zones, particulièrement bondés et exposés à la chaleur estivale, pourront devenir des lieux propices aux situations stressantes et, par conséquent, accroître le risque d’arrêt cardiaque. En France, plus de 40 000 personnes font face à cette situation chaque année, avec un taux de survie de seulement 6 %. Le manque de formation aux gestes qui sauvent persiste et la majorité des victimes succombent dans les dix minutes qui précèdent l’arrivée des secours. Par comparaison, la Suède affiche un taux de survie de 40 %, principalement grâce à une population largement formée aux premiers secours, à un accès aisé aux défibrillateurs et à un entretien méticuleux Malgré des progrès ces dernières années, notre pays accuse un retard significatif dans ce domaine : les défibrillateurs automatisés externes (DAE) sont mal entretenus et insuffisamment déclarés aux associations de citoyens sauveteurs. De plus, la fermeture d’établissements équipés de DAE rend ces équipements médicaux parfois inaccessibles, alors que le nombre de citoyens capables d’administrer les premiers secours demeure faible. Madame la ministre, à l’approche des Jeux, Jeux, je vous interpelle sur les mesures concrètes que le Gouvernement envisage de prendre pour assurer la protection des spectateurs et des visiteurs contre le risque d’arrêt cardiaque. Plus généralement, comment comptez vous renforcer

La loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque a imposé l’obligation d’équipement en DAE des établissements recevant du public public (ERP), le renforcement de la signalétique relative à ces équipements, leur maintenance et, enfin, la création d’une base de données nationale Géo’DAE pour les recenser et, surtout, les géolocaliser. L’enjeu est d’améliorer les chances de survie en permettant à une personne témoin d’un arrêt cardiaque de disposer très rapidement d’un DAE en complément de la réalisation des gestes de premiers secours. La déclaration des informations relatives à ces dispositifs médicaux par leurs propriétaires ou par les professionnels assurant la maintenance des DAE sur le portail Géo’DAE intervient dans le respect du standard défini par l’arrêté du 29 octobre 2019 Elle a pour objectif de faciliter leur géolocalisation par les services de secours et d’aide médicale urgente, ainsi que par des applications citoyennes diffusant les données relatives aux DAE. Depuis la création de la base de données nationale au mois de mars 2020, on observe une augmentation croissante du nombre de déclarations. En effet, près de 112 000 DAE ont ainsi été déclarés.

Elles permettent aussi à certaines applications disponibles sur les différentes plateformes de mobiliser des citoyens sauveteurs en cas d’arrêt cardiaque tout en géolocalisant les DAE et, ainsi, de sauver des vies. Des actions de sensibilisation et de communication sont régulièrement assurées pour améliorer la déclaration des données relatives aux DAE installés et, ainsi, contribuer au déploiement de la base nationale Géo’DAE. Des QR codes DAE ont été placés dans des endroits stratégiques des territoires pour maximiser la visibilité et l’accessibilité de ces instruments pour le grand public afin de les intégrer au mieux dans la chaîne de prise en charge de l’arrêt cardiaque.

en 2018, le Gouvernement a, par ordonnance, clarifié les dispositions relatives aux conditions d’autorisation d’ouverture des officines de pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants, par voie de création, de transfert ou de regroupement. Ce texte a prévu des dispositions en faveur des territoires au sein desquels l’accès au médicament pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante. Les critères d’éligibilité de ces territoires devaient être définis par décret.

Nous voilà en janvier 2024. Qu’en est il, madame la ministre ? Vous semble t il normal que les parlementaires, comme l’ensemble des élus du territoire, aient l’impression que l’on se moque d’eux ? La parole est

Le code de la santé publique prévoit, en effet, qu’un décret doit déterminer les conditions de définition des territoires au sein desquels l’accès au médicament pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante. Le maillage officinal est aujourd’hui globalement satisfaisant : au 1 janvier 2023, on comptait 20 142 officines sur l’ensemble du territoire, ce qui correspond à trente officines pour 100 000 habitants. Au sein des territoires identifiés comme fragiles, le maillage des officines pourra être renforcé grâce à des aides financières en vue de favoriser le maintien ou l’installation d’une officine ou grâce à un assouplissement des règles encadrant les autorisations de transfert et de regroupement. Cet aménagement contribuera notamment au renforcement du maillage des officines dans les communes de moins de 2 500 habitants, car elles auront la possibilité d’être regroupées avec des communes contiguës afin qu’une officine soit autorisée à y ouvrir.

je veux vous assurer de la détermination de la ministre du travail, de la santé et des solidarités à publier le plus rapidement possible ces textes, une fois que celles ci seront terminées. les agences régionales de santé (ARS) pour réaliser un point d’étape sur la rédaction de ce décret. L’objectif partagé est d’aboutir à une méthodologie plus claire et plus adaptée aux enjeux du maillage officinal.

30 % des capacités d’hospitalisation de ces deux hôpitaux, l’hôpital Bichat et l’hôpital Beaujon, qui seraient purement et simplement rayées de la carte. Ce projet est d’autant plus inquiétant qu’il se situe dans le nord est parisien, dans une des zones les plus carencées d’Île de France : on y compte

Il offrira des conditions d’accueil pour les patients et d’exercice pour les professionnels de santé sans commune mesure avec ce qu’elles sont aujourd’hui à Bichat et Beaujon.

Ce projet permettra de rééquilibrer géographiquement l’offre de maternité en faveur de la Seine Saint Denis, sans déstabiliser l’offre de soins du territoire. Dans tous les cas, l’implantation de ce nouvel établissement ne déstabiliserait pas l’offre de soins en maternité, puisque les autres maternités du territoire seraient capables d’absorber le solde des naissances.

Pour toutes les questions relevant de la déclaration d’utilité publique, le ministère du travail, de la santé et des solidarités a bien entendu connaissance des démarches judiciaires en cours et les suit avec attention.

et numérique. Madame la ministre, à l’heure où l’énergie n’a plus de ministère de plein exercice et où le projet de loi sur la souveraineté énergétique ne donne malheureusement aucune visibilité de volume pour les énergies renouvelables, il est plus que jamais nécessaire de s’interroger sur le soutien de l’État à la filière hydrolienne et sur la traduction des annonces du Président de la République aux Assises de l’économie de la mer, à Nantes, le 28 novembre dernier. Si le Gouvernement souhaite une relance forte du nucléaire, les nouvelles capacités nucléaires ne seront pas connectées avant 2035. En parallèle du soutien à la filière électronucléaire et en vue de pleinement décarboner le mix énergétique, il est indispensable d’accélérer dès à présent le développement massif des énergies renouvelables, notamment marines, comme le recommande le rapport de RTE (Réseau de transport d’électricité). Après l’échec d’OpenHydro en 2018, faute d’un soutien clair et franc de l’État à la filière, l’annonce du soutien financier à hauteur de 65 millions d’euros à la ferme pilote hydrolienne manchoise FloWatt était inespérée. En effet, l’énergie hydrolienne était encore laissée pour compte dans le cadre de la précédente programmation pluriannuelle de l’énergie malgré les deux courants puissants et très prometteurs que l’on rencontre au raz Blanchard, à la pointe du Cotentin, et dans le passage du Fromveur, dans le Finistère. La stratégie de développement de la filière hydrolienne repose sur la nécessaire visibilité de développement commercial à court terme, condition indispensable aux investissements, donc à la baisse des coûts de cette nouvelle filière industrielle française prometteuse. Il s’agirait pour l’État de lancer dès à présent des appels d’offres commerciaux, sans attendre les mises en service des fermes pilotes. C’est d’ailleurs ainsi qu’a été appréhendé le développement de l’éolien flottant. Attendre serait néfaste pour l’ensemble de la filière et pour la société HydroQuest elle même, à l’origine de FloWatt. effet, cela impliquerait une possible rupture d’activité et de charge de plusieurs années entre le moment de la livraison des hydroliennes de la ferme pilote en 2026 et le moment où la société serait susceptible d’être lauréate d’un projet commercial en France. Ces défis et les difficultés rencontrées par la filière hydrolienne n’ont pas empêché la Grande Bretagne de la développer de manière extrêmement volontariste. Madame la ministre, le Gouvernement va t il s’engager à lancer rapidement des appels d’offres commerciaux, afin que la filière industrielle française de l’hydrolien devienne enfin une réalité ? La parole est à Mme la ministre Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui, ne pouvant être présent ce matin, m’a chargée de vous répondre. Les différentes sources d’énergies renouvelables sont complémentaires et ont vocation à contribuer, chacune selon son potentiel, à l’atteinte de nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique et de souveraineté énergétique. À ce titre, les nouvelles énergies marines présentent un potentiel que nous intégrons pleinement dans nos réflexions sur notre prochaine stratégie énergétique. La France a été pionnière dans l’exploitation de l’énergie des marées, avec l’usine marémotrice de la Rance, de la Rance, première installation au monde à produire de l’électricité à partir de l’énergie des marées à une échelle industrielle. Cependant, une telle installation présente aussi des inconvénients, par exemple l’ensablement progressif de la Rance, qui nécessite des interventions et des travaux réguliers. La stratégie de la Commission européenne, publiée au mois de novembre 2020 a fixé l’objectif de 40 gigawatts de capacité d’énergie océanique hors éolien en mer et de 300 gigawatts d’éolien en mer dans l’Union européenne d’ici à 2050. Concernant l’hydrolien en mer, la France, par ses courants marins, notamment ceux du raz Blanchard et du passage de Fromveur, présenterait un potentiel maximum estimé entre 3 et 5 gigawatts. Pour autant, par rapport à d’autres énergies comme le solaire ou l’éolien terrestre et en mer, cette technologie reste à un stade de développement amont et doit encore poursuivre sa montée en maturité, en particulier afin de réduire ses coûts par rapport à d’autres énergies renouvelables.

Dans cette perspective, le Gouvernement travaille actuellement pour que la prochaine politique pluriannuelle de l’énergie intègre le lancement de premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, sous réserve d’une baisse des coûts de la technologie.

par des difficultés d’accès à des dispositifs d’aide et d’accompagnement à la rénovation énergétique mis en place par l’État, rénovation énergétique elle même évidemment indispensable face aux changements climatiques.

de vous répondre. Le chauffage domestique au bois constitue, d’une part, l’une des principales sources actuelles de chaleur renouvelable, d’autre part, la principale source d’émissions de particules fines.

est en cours de déploiement depuis la fin de 2021. Les aides au renouvellement des appareils de chauffage au bois déployées à l’échelon national sont maintenues en 2024.

Il est primordial que MaPrimeRénov’ puisse continuer à soutenir l’installation d’appareils très performants de chauffage aux granulés ou au bois. Cela permet de décarboner les bâtiments en remplaçant les équipements fioul ou gaz sans impact pour le système électrique. Sous l’impulsion de la politique du Gouvernement, le marché des chaudières biomasse est passé de 10 000 chaudières par an en 2018 à 42 000 en 2022. Cela permet de réduire les émissions de particules grâce au remplacement d’appareils existants alimentés à la biomasse.